La séance est reprise. L'ordre du jour appelle la désignation des vingt et un membres de la commission d'enquête sur les réponses apportées par les autorités publiques au développement de la radicalisation islamiste et les moyens de la combattre. En application de l'article 8 , alinéa 5 de notre règlement, les listes des candidats présentés par les groupes ont été publiées. Ces candidatures seront ratifiées si la présidence ne reçoit pas d'opposition dans le délai d'une heure prévu par notre règlement. Mes chers collègues, j'ai le plaisir de saluer la présence dans la tribune d'honneur d'une délégation du Conseil fédéral d'Autriche, conduite cet après-midi par son vice-président, M. Hubert Koller. La délégation est accompagnée par notre collègue François Bonhomme, président du groupe interparlementaire d'amitié. Elle a été reçue ce matin en audience par le président Gérard Larcher, en présence de M. Karl Bader, président du Conseil fédéral d'Autriche. Elle a ensuite échangé avec notre collègue questeur Rémy Pointereau sur la thématique des zones de revitalisation rurale, puis elle s'est entretenue avec les membres du groupe interparlementaire d'amitié France-Autriche. Formons le voeu que cette visite en France contribue à renforcer encore les liens historiques qui unissent nos deux assemblées et nos deux pays. Mes chers collègues, en votre nom à tous et au nom du Sénat, permettez-moi de souhaiter à nos homologues du Conseil fédéral d'Autriche la plus cordiale bienvenue, ainsi qu'un excellent et fructueux séjour.

Nous proposons, par cet amendement, d'instaurer un malus sur les cotisations patronales dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les entreprises présentant une sinistralité anormalement élevée.

ces chiffres ne prennent pas en compte les milliers d'accidents non déclarés à la sécurité sociale et les milliers de salariés victimes de maladies professionnelles non reconnues comme telles. Il est temps de faire prendre aux employeurs une autre direction que celle qu'ils continuent de suivre en refusant d'engager les dépenses nécessaires à la protection de la santé et de la sécurité de leurs salariés. C'est un sujet beaucoup trop important pour qu'il ne fasse pas partie des priorités en matière de gestion du personnel. Il est inacceptable en effet que, aujourd'hui, les salariés prennent des risques au travail physique et mentale. Il est d'ailleurs très malheureux que le Gouvernement ait décidé, dans les ordonnances « Travail », de supprimer les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, institutions qui jouaient un rôle majeur dans la prévention des risques professionnels, et qu'il s'apprête à réformer dans le mauvais sens les services de santé au travail. C'est pourquoi nous proposons de renforcer les sanctions à l'égard des entreprises qui sont à la traîne en matière de sécurité au travail et de relever les taux de cotisations auprès de la branche AT-MP des entreprises présentant une sinistralité anormalement élevée. Cette tarification des risques professionnels permettrait de dégager des fonds nécessaires pour la réparation, l'évaluation et la prévention des risques professionnels et participerait ainsi à la promotion de la santé au travail. La parole est

grâce à un mécanisme de malus pour les employeurs n'ayant pas pris les mesures nécessaires pour éliminer le risque avéré d'épuisement professionnel. Dans leur rapport d'information du 15 février 2017 relatif au

il est prévu de relever les taux de cotisations auprès de la branche AT-MP des entreprises présentant une sinistralité anormalement élevée. Cette tarification des risques professionnels permettrait de dégager des fonds pour la réparation, l'évaluation et la prévention des risques professionnels, et participerait à la promotion de la santé au travail.

Certains secteurs présentent aussi un taux de sinistralité anormalement élevé, au premier rang desquels celui de l'intérim, suivi par celui de l'aide et des soins à la personne. La hausse de la part liée à la sinistralité dans le calcul du taux mixte de cotisation n'est pas étrangère à cette évolution globale favorable à la sinistralité. C'est pourquoi nous souhaitons renforcer la responsabilisation financière des entreprises, en leur imputant une part plus significative- deux tiers -du coût des accidents du travail et des maladies professionnelles, quels qu'ils soient. Quel est l'avis de commission ? Cet amendement tend à revenir sur l'équilibre actuel des responsabilités entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice, en reportant sur cette dernière la plus grande partie de la responsabilité. Or il ne faut pas oublier que l'entreprise de travail temporaire demeure aujourd'hui responsable de la médecine du travail des salariés intérimaires, notamment de leur formation à la prévention et au respect des exigences de sécurité. Une révision des modalités de tarification des AT-MP requiert donc au préalable une réévaluation de la répartition des responsabilités

de déclaration d'emplois ponctuels pour les associations, ainsi que pour les organismes permanents à caractère social des collectivités locales et des entreprises qui auraient recours à de tels emplois dans le cadre de manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées, dans l'année, à leur profit exclusif. En effet, lors de manifestations de ce type, et pour une question de logistique, il est fréquemment fait appel à des emplois ponctuels, le plus souvent pour quelques heures seulement, afin de sécuriser un parking, tenir des toilettes, etc. Aujourd'hui, l'Urssaf impose aux représentants des associations et des organismes permanents à caractère social des collectivités locales et des entreprises de réaliser des déclarations pour chacun de ces emplois, même pour quelques heures de poste, sous peine de sanctions, alors même que ces emplois répondent, dans leur grande majorité, aux critères de réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires. Il ne s'agit donc pas tant, en particulier pour les associations, de réduire les coûts, mais bien de répondre aux difficultés engendrées par une tâche particulièrement chronophage pour les gestionnaires qui sont le plus souvent des bénévoles. Dans un souci de simplification, cet amendement vise à exclure de la liste de l'assiette de la contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement ces emplois ponctuels, uniquement au bénéfice des associations

Par ailleurs, la proposition nous paraît introduire une forme de confusion entre des situations différentes : d'un côté, la situation du personnel bénévole, qui s'engage de manière libre et gratuite, de l'autre, celle du personnel salarié, qui s'engage contre une rémunération, laquelle, à nos yeux, doit être réglementée et contrôlée. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons être que défavorables à cet amendement, même s'il existe encore- j'en suis sûr -des marges de progrès en matière de simplification. Soyez d'ailleurs assuré que nous nous attachons

est à M. le secrétaire d'État. Je ne veux pas laisser traduire mes propos dans un sens qui ne serait pas exact : je n'ai pas dit que les associations recouraient au travail dissimulé, j'ai dit que l'application de cet amendement reviendrait à traiter la rémunération des personnels concernés comme celle

pour la pratique d'activités physiques et sportives en entreprise. Cette mesure est préconisée de longue date par les partenaires sociaux, par les représentants patronaux et par différents rapports. Il s'agit également d'une annonce faite par le Premier ministre à l'occasion d'un comité interministériel pour les jeux

Ainsi, les prestations en nature ou en espèces liées à des activités sociales et culturelles servies par les comités d'entreprise sont exonérées de cotisations. De ce fait, la plupart des aides à l'activité sportive délivrées par le comité social et économique d'une entreprise ou par l'employeur, en l'absence de comité, sont exonérées. Pour permettre le développement de la pratique du sport en entreprise, des travaux complémentaires sont en cours- ils ont été cités -afin de clarifier les critères d'exonération des avantages liés aux activités sportives, notamment en ce qui concerne la mise à disposition de locaux.

Depuis le 1 avril 2013, l'ASPA est égale à 787,26 euros par mois pour une personne seule et à 1 222,27 euros pour un couple. Cette allocation relève de la solidarité nationale, conformément au préambule de la Constitution de 1946, selon lequel la Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. Aujourd'hui, de nombreuses personnes âgées qui pourraient être bénéficiaires de l'ASPA refusent de faire valoir leurs droits du fait du prélèvement sur succession qui aura lieu après leur décès pour rembourser l'allocation octroyée. Ce système doit être modifié. Alors que nous luttons contre le non-recours, les familles ne doivent pas renoncer à un droit par peur que leurs enfants ou petits-enfants

Pour rétablir la solidarité nationale, nous proposons de supprimer le dispositif de remboursement sur succession. Quel anciennement appelé minimum vieillesse, relève d'une logique non contributive de solidarité nationale. Elle assure à la personne âgée ou invalide un complément de revenu qui s'agrège à la pension afin que ses revenus atteignent un niveau minimum. C'est en vertu de cette logique non contributive qu'elle est récupérable sur succession après le décès du bénéficiaire. Elle se substitue en quelque sorte à l'obligation de solidarité familiale. De plus, l'assiette de la récupération a plusieurs fois été modifiée

rapporteur général. Cet amendement a pour objet d'augmenter provisoirement le taux de la taxe de solidarité additionnelle (TSA) due par les organismes complémentaires d'assurance maladie. En effet, ces organismes font part de plus en plus ouvertement de leur intention d'augmenter leurs tarifs au fur et à mesure de l'application du reste à charge zéro- c'était ce que nous craignions,

et contreviendrait totalement à l'esprit du dispositif adopté dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019. Face à cela, cet amendement tend à proposer une mesure conservatoire.

organismes complémentaires qui appartiennent à de grands groupes et qui versent des dividendes à des actionnaires.

après les interventions de l'assurance maladie et de l'assurance complémentaire. À ce jour, les complémentaires santé ont pour seule obligation, dans le cadre des contrats responsables, de pratiquer le tiers payant sur le ticket modérateur. À titre d'illustration, cela ne représente que 12 % de la dépense sur un panier 100 % santé en optique. Alors que cette offre doit permettre de lutter contre toutes les formes de renoncement aux soins pour des raisons financières, sa pleine et entière appropriation par les Français ne pourra être effective que s'ils sont assurés d'être à la fois intégralement remboursés et de ne pas avoir à faire d'avance de frais.

prévoyons également qu'un organisme complémentaire qui ne mettrait pas en oeuvre l'accès à un tiers payant intégral sur le forfait perde l'avantage fiscal dont il bénéficie au titre du contrat responsable.

En complément de la réforme du reste à charge zéro pour l'optique et les prothèses dentaires et auditives adoptée l'année dernière, cet amendement vise à restreindre les pratiques de différenciation des remboursements de certains organismes complémentaires selon que les assurés ont eu recours ou non à des professionnels partenaires d'un réseau de soins. La mise en place du 100 % santé au 1 janvier 2020 va recentrer ces réseaux sur les offres du marché libre, pour lesquelles les remboursements de l'assurance maladie obligatoire seront, en ce qui concerne l'optique, fortement diminués. Ainsi, avec cet amendement, nous voulons éviter que les assurés qui décideraient, par exemple, de ne pas avoir recours au panier 100 % santé sans reste à charge puissent se voir appliquer des remboursements différenciés, au-delà d'un seuil fixé par décret, par leur organisme complémentaire. Les contrats qui prévoiraient des clauses de ce type ne seraient pas éligibles au taux réduit de taxe de solidarité additionnelle applicable aux contrats responsables et solidaires. Cet amendement s'inscrit dans une logique d'équité entre les assurés, à cotisation égale, et vise à défendre leur liberté de choisir leurs professionnels de santé. il permettrait d'éviter les abus en la matière. de reste à charge, le présent amendement vise à encadrer la pratique du remboursement différencié. En effet, cette pratique permet actuellement aux complémentaires de moins bien rembourser leurs assurés qui ne se rendraient pas chez un professionnel de santé affilié à leur réseau de soins, y compris lorsque ces assurés se rendent Alors que de nombreux territoires ne disposent pas de professionnels affiliés à ces réseaux, le remboursement différencié peut aggraver les inégalités territoriales d'accès

amendements identiques d'accélérer le déploiement du tiers payant intégral sur les offres de reste à charge zéro.

d'un tiers payant intégral, qui pourra être généralisable à tous les assurés dans des conditions techniques fiabilisées, sans toutefois l'imposer. Les échanges sont engagés depuis plusieurs années avec les organismes complémentaires, la récente loi qui permet la résiliation à tout moment des contrats de complémentaire santé a par ailleurs mis en place un suivi de la mise en oeuvre des outils numériques permettant à ces organismes d'assurer le tiers payant.

visent à prévenir des pratiques de remboursement différenciées par les organismes complémentaires d'assurance maladie selon que les patients ont recours ou non à un professionnel de santé adhérent à un réseau de soins.

contient, selon nous, les prémices de votre projet de mettre fin à notre système de retraite par répartition. En effet, comme l'étude d'impact du projet de loi le précise, « ces différentes étapes permettront que l'unification du recouvrement des cotisations sociales constitue utilement un acquis pour la mise en oeuvre future de la réforme des retraites. » Est-ce ainsi que le Gouvernement entend procéder désormais, c'est-à-dire en anticipant la mise en oeuvre technique d'une réforme qui n'a pas encore été adoptée ? Cela montre que vous faites fi de la pseudo-concertation engagée avec les organisations syndicales sur votre réforme.

Même si l'oeuvre d'unification est effectivement en cours depuis 2011, elle interroge sur l'autonomie de gestion des organismes, qui ne recouvrent pas tous le même type de contributions et de cotisations.

À ce sujet, l'une des dispositions de cet article met en cause l'autonomie de gestion de l'Unédic, pourtant garantie jusqu'à présent dans la convention quadripartite conclue notamment entre l'Unédic, Pôle emploi et l'Agence

commission ? L'avis est défavorable, par cohérence avec la position de la commission, qui préconise justement l'adoption de cet article. L'unification du recouvrement dans la sphère sociale présente de réels défis, mais, si elle est bien menée,

C'est aussi un avis défavorable. Avec cet article, nous avons la volonté de mettre en oeuvre les préconisations du rapport de M. Alexandre Gardette, remis en septembre dernier au Gouvernement sur l'unification du recouvrement dans les sphères sociales et fiscales, avec des objectifs de simplification pour les employeurs et les entreprises,

qu'en est-il des régimes de retraite complémentaires, gérés notamment par la Caisse des dépôts et consignations ? Qu'en est-il des régimes de retraite de l'État,

le secteur privé ? Comment voyez-vous les choses, monsieur le secrétaire d'État ? Ne pensez-vous pas qu'il eût été intéressant, pour entraîner ce mouvement vers la performance, que l'État soit le premier à montrer l'exemple ?

; il concerne également le régime de la fonction publique et les régimes spéciaux, à l'exception des plus petits d'entre eux, qui n'ont qu'un employeur, pour lesquels nous ne voyons pas d'utilité particulière à procéder à un tel regroupement.

Nous proposons au Parlement un certain nombre de dispositions dans cet article 10. Nous avons en revanche retiré du projet initial que nous avions imaginé un certain nombre d'autres dispositions, que vous avez citées, car il nous a semblé, après échanges,

Vous proposez pour les entreprises éphémères de substituer à la DSN plusieurs déclarations auprès des différents organismes auxquels est normalement adressée la DSN. Cela ne nous paraît pas nécessairement être le meilleur moyen de lutter contre la fraude. Nous considérons en effet que les entreprises éphémères

nous pensons utiliser vos travaux pour orienter la politique de contrôle des organes compétents sur les entreprises qui relèvent de critères identifiés, notamment les entreprises éphémères, dont vous avez démontré

Toutefois, le projet de loi ne vise expressément que les cotisations du régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales, les cotisations des régimes d'assurance vieillesse complémentaire et invalidité-décès, omettant de faire référence aux cotisations du régime des prestations complémentaires de vieillesse des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, également recouvrées par les caisses de professions libérales. Par ailleurs, l'alinéa 18 de l'article dresse la liste des cotisations recouvrées par les Urssaf, notamment dans le cadre du régime simplifié des professions médicales (RSPM) pour les médecins remplaçants et étudiants

les cotisations des régimes complémentaires et invalidité-décès, ainsi que la cotisation d'ajustement du régime de prestations complémentaires de vieillesse des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, omettant lui aussi de faire référence à la cotisation proportionnelle de ce dernier régime, applicable aux médecins relevant du RSPM, introduite par l'article 36 du présent projet de loi. Il vise par erreur l'article L. 645-1, qui ne mentionne quant à lui aucune cotisation. Le présent amendement vise par conséquent à rectifier ces différentes erreurs et omissions.

Sur le principe, la commission est favorable à la démarche d'unification, gage d'efficacité et de simplicité pour les usagers.

pour le préjudice présentant un caractère anormal et spécial. Le préjudice devrait être pris en charge par l'Acoss, car cette mesure s'inscrit dans le contexte global de la restructuration et de l'unification du recouvrement de la sphère sociale. Notre amendement a pour objet de sécuriser juridiquement le principe de prise en charge de l'indemnisation par l'Acoss plutôt que par l'État.

le régime microsocial, vous le savez, prévoit en particulier une procédure d'enregistrement simplifiée et offre une meilleure lisibilité des cotisations sociales qui sont indexées sur le chiffre d'affaires et payées mensuellement ou trimestriellement. Ce régime n'était pas en vigueur à Mayotte, alors même que ce territoire de notre pays, la France, est un département depuis 2011. La transposition du régime microsocial aurait pourtant participé à la création d'emplois et au développement économique du territoire. Cette extension aurait également concouru à la lutte contre certaines pratiques informelles. Elle aurait répondu à une demande forte des organismes créateurs d'activité économique, tels que l'Association pour le droit à l'initiative économique (ADIE). C'est la raison pour laquelle j'avais, en 2017, lors de l'examen du projet de loi de programmation relative à déposé un amendement visant à rendre effectif dans le département de Mayotte le régime microsocial, adopté, vous le savez, en 2008 dans le cadre de la loi de modernisation de l'économie et renforcé en 2014 dans la loi relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises. La commission des affaires sociales et le Gouvernement m'avaient à l'époque demandé de le retirer, car, selon eux, une extension du régime microsocial à Mayotte était difficilement envisageable à la date de promulgation de la loi, dans la mesure où il ne pouvait être transposé tel quel. Il fallait prendre le temps nécessaire à sa mise en oeuvre. Je suis donc ravi aujourd'hui que l'article 11 prévoie enfin d'étendre au département de Mayotte le régime microsocial, l'allégement des démarches afférentes aux charges sociales et à l'impôt sur le revenu pour les petites entreprises. Les acteurs locaux qui se sont battus pour ce résultat, au premier rang desquels l'ADIE, doivent donc être félicités

il n'est pas nouveau.

hôteliers, gîtes ruraux, etc. Des réponses partielles ont été apportées par l'article 18 de la loi du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, qui prévoit l'assujettissement des loueurs aux cotisations sociales, l'article 44 de la loi du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, qui prévoit l'obligation pour les plateformes de collecter la taxe de séjour, et par l'article 10 de la loi du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude, transmission automatique des revenus des utilisateurs des plateformes à l'administration fiscale. Si le principe de l'assujettissement aux cotisations sociales des loueurs en meublés de tourisme a été entériné, son application pratique pose question, les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale ayant été laissées à l'écart des récents mécanismes de transmission automatique des revenus. Le seuil retenu pour l'assujettissement des loueurs a été fixé à 23 000 euros par an. Les loueurs de biens dits « meubles »- voitures, tondeuses -sont assujettis aux cotisations sociales dès le dépassement du seuil de 20 % du plafond de la sécurité sociale, soit 8 104,80 euros en 2019. Il y a donc deux catégories de loueurs, selon le type de bien loué. Par ailleurs, un loueur mettant à disposition sa résidence principale jusqu'au seuil maximum de 120 jours par an à un prix moyen de 80 euros la nuit gagne au maximum 9 600 euros par an. Tous les revenus tirés de son activité de location sont donc exonérés de cotisations sociales. L'objet de cet amendement est d'aligner le régime de cotisation des loueurs de meublés sur celui des biens meubles. Un nombre important de loueurs de meublés demeureront non assujettis puisque, selon la plateforme Airbnb, le revenu moyen annuel des hébergeurs est d'environ 2 000 euros.

pour adopter une telle disposition. Par ailleurs, sur la forme, je partage totalement l'avis du rapporteur général sur un rattachement au code général des impôts plutôt qu'à un projet de loi

Le principe est similaire au texte voté dans la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude. Les plateformes de mise en relation deviendraient tiers déclarant, comme peuvent déjà l'être aujourd'hui les associations et centres de gestion ou les cabinets d'expertise comptable, la déclaration sociale nominative. Elles seraient aussi responsables du versement des cotisations et contributions sociales. Cette mesure faciliterait le contrôle de l'activité de location de locaux d'habitation meublés à titre lucratif, la lutte contre la fraude, l'acquisition de droits à prestations de sécurité sociale par les loueurs. Par cohérence, le code général des impôts est amendé pour contraindre les plateformes à informer l'administration sociale dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour l'administration. Je m'attends à votre réponse, monsieur D'une part, il tend à inclure les loueurs de meublés de vacances dépassant le seuil de 23 000 euros de chiffre d'affaires par an dans le dispositif- c'est aujourd'hui optionnel -par lequel les entrepreneurs indépendants peuvent autoriser les plateformes à effectuer pour eux leurs déclarations. Cela me paraît une excellente chose.

et le dispositif pourra sans doute être revu, mais il sera intéressant d'entendre le Gouvernement sur ses intentions dans l'immédiat ou à l'avenir.

Aussi, l'assimilation à la DSN que vous proposez ne nous paraît pas tout à fait opportune. Pour les indépendants, l'article L. 613-6 du code de la sécurité sociale permet déjà aux plateformes de jouer le rôle de tiers déclarant lorsque les particuliers exercent l'activité en tant qu'auto-entrepreneurs.

administrative de la prise en charge des services d'aide à domicile ou d'aide à la personne. Cet article permettra d'alléger le casse-tête que peut parfois représenter

Pour les familles, pour les salariés, un cadrage national ne peut évidemment être qu'un mieux. Tirons donc les enseignements de ces expérimentations afin d'évoluer vers un statut des aides à domicile et un plancher de rémunération. L'étude nationale des coûts avait établi le prix rémunérateur à 25 euros de l'heure en moyenne. Or nous sommes trop souvent en deçà de ce tarif, ce qui entraîne une compression des coûts pour les structures ou un reste à charge important pour les familles. La parole

est tout sauf un cadeau aux services d'aide à domicile. Cette mesure est réservée aux particuliers employeurs résidant à leur domicile et aux usagers de certains prestataires d'aide à domicile, au titre des services à la personne

En d'autres termes, la contemporanéité soutient la demande, à une nuance près, puisqu'il a été démontré que le crédit d'impôt bénéficie avant tout au 1 % des Français les plus aisés.

secteur des salaires corrects et de véritables parcours de formation, mettre en oeuvre des pratiques de direction innovantes et respectueuses de la personne humaine. Des conditions de travail suffisamment attractives

L'article 13 poursuit la logique entamée l'année dernière de gradation des sanctions en fonction de la gravité du manquement constaté. Actuellement, les sanctions applicables en matière de travail dissimulé sont les mêmes pour tous les employeurs, indépendamment de la taille de l'entreprise ou de la gravité des infractions constatées. Elles se traduisent par une annulation des exonérations de cotisations sociales. La tendance est à l'affaiblissement des sanctions en cas de travail illégal, notamment. Le fait de dissimuler le travail de plusieurs personnes ou de commettre une infraction de travail dissimulé en bande organisée ne constituera plus une circonstance

Alors que votre gouvernement a lancé une chasse implacable contre les fraudeurs aux prestations sociales, les sanctions appliquées aux entreprises en cas de fraude à la sécurité sociale se verraient amoindries. Pour nous, il y a véritablement deux poids, deux mesures

tous les employeurs, indépendamment de la taille de l'entreprise ou de la gravité des infractions constatées, se traduisent par une annulation des exonérations de cotisations sociales.

la fraude fiscale est très certainement plus importante que la fraude sociale. Merci de le reconnaître ! Ce n'est pas parce que l'une est plus importante que l'autre qu'il ne faut pas combattre les deux. Je suis, en les deux. Je suis, en revanche, en désaccord avec vous lorsque vous dites qu'on donne un blanc-seing à la fraude fiscale des entreprises. Ce gouvernement a fait adopter la loi du 23 octobre 2018 qui renforce les moyens de lutte contre la fraude. Pour vous donner une seule illustration, l'année 2019 sera une

au renforcement de la lutte contre la fraude sociale qui, en plus de desservir les intérêts des travailleurs, gangrène le budget de la sécurité sociale. À cet égard, les arguments de notre collègue Fabien Gay devraient faire réfléchir chacune et chacun d'entre nous. nous sommes déjà largement expliqués sur ce sujet. La lutte contre la fraude passe aussi par l'arrêt des suppressions de postes d'inspecteurs du travail, par le recrutement massif d'agents et par l'harmonisation vers le haut des droits sociaux

Comment les agents de contrôle pourraient-ils remplir convenablement leurs missions quand l'objectif est de réduire toujours plus les effectifs ? S'agissant de la politique de la France en matière de travail détaché,

Vous pouvez essayer de minimiser ce montant, il n'en reste pas moins que ces dizaines de milliards d'euros devraient constituer la principale cible du Gouvernement pour accroître les ressources de la sécurité sociale.

des retraités français établis hors de France de percevoir leurs pensions sur un compte domicilié à l'étranger et les obligerait à détenir un compte domicilié en France pour ensuite organiser le transfert des fonds. Cette mesure constitue une forme de punition collective, si vous me permettez cette comparaison. C'est la raison pour laquelle nous vous demandons de retirer votre amendement,

que des annonces concrètes devraient être faites dans les heures ou les jours à venir. Il s'agit là d'un mépris total pour le travail parlementaire. Je tiens à le dénoncer et je m'associe à la demande de mes collègues de suspendre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

La séance est reprise. Monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, je vais de nouveau suspendre la séance. Je vous informe que M. le président du Sénat

La séance est reprise. Mes chers collègues, la conférence des présidents réunie ce jour a décidé de poursuivre l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 afin de permettre au Sénat de se prononcer sur la troisième partie et sur l'ensemble du texte ce soir même. En conséquence, le vote solennel du mardi 19 novembre est annulé. La conférence des présidents a également décidé, en accord avec le Gouvernement, d'inscrire la nouvelle lecture du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 à l'ordre du jour du samedi 30 novembre et du dimanche 1 décembre matin, midi et soir. Le délai limite pour le dépôt des amendements de séance pourrait être fixé au jeudi 28 novembre à midi. L'ordre du jour résultant de ces modifications sera mis en ligne sur le site du Sénat.

corps intermédiaires, s'il veut encore une fois « uberiser » ou désintermédier la politique, il risque de connaître un grave désenchantement et d'accroître les tensions dans un climat social qui est aujourd'hui explosif. Oui, vous prenez le risque

qui existent précisément pour que le climat, au moins politique, reste serein et que l'on puisse engager une conversation civique, quelles que soient les positions des uns et des autres, sur des bases sincères.

On a lu beaucoup de choses dans la presse. Que le Président de la République prenne la mesure du problème hospitalier, c'est une bonne chose, et on ne peut que s'en réjouir, mais le problème est connu, il n'est pas nouveau. Pourquoi les mesures annoncées ne figuraient-elles pas dans le projet de loi de financement qui nous a été soumis ?

contre les politiques d'austérité qui sont menées depuis des décennies dans le secteur de la santé, et qui ont fortement détérioré les conditions de prise en charge

ces quinze dernières années. Cet après-midi, alors que la manifestation n'était pas terminée et que nous débattions ici de l'article

présentée au début des travaux sur le PLFSS. Ce n'est pas acceptable vis-à-vis des parlementaires, lesquels se sont beaucoup investis sur le texte,

Pour toutes ces raisons, le groupe CRCE souscrit aux conclusions de la conférence des présidents et n'adoptera pas la partie relative aux recettes de ce PLFSS.

Oui, l'hôpital est malade, et cela ne remonte pas à la semaine dernière ! Ce n'est pas une urgence ; c'est une maladie chronique qui s'est acutisée, pour employer des termes médicaux.

Non, la démocratie ne peut pas se résumer à un dialogue direct entre la rue et le Président de la République, par l'intermédiaire des chaînes d'information en continu, et ce au mépris de tous les corps intermédiaires,

dans des circonstances qui sont, je le répète, exceptionnelles. Il est normal que le Président de la République s'exprime le jour où un mouvement social d'importance est en cours dans notre pays.

auquel nous travaillons encore à cette heure : dégager des moyens financiers pour l'hôpital ; élaborer un grand plan d'attractivité pour répondre aux difficultés de recrutement, qui sont l'une des principales sources du mal-être des soignants

Les mesures relevant de la loi seront, comme je vous l'ai déjà garanti, inscrites dans le PLFSS en nouvelle lecture, ce qui ne privera le Parlement ni d'une discussion ni d'un vote. Je prends acte ce soir de votre décision de ne pas poursuivre le débat. Je le regrette, car les mesures en dépenses qui vous sont proposées par le Gouvernement me semblaient mériter d'être discutées.

J'entends parler d'instrumentalisation du Parlement, de mise en cause de la crédibilité de la parole gouvernementale ou de celle des institutions parlementaires. Cette analyse me paraît quelque peu exagérée. Il arrive, et c'est le cas dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, que le calendrier politique et le calendrier parlementaire entrent en collision ou, du moins, ne suivent pas le même rythme. C'est l'essence même de la politique que de faire face à l'imprévu

Deux solutions ont été examinées en conférence des présidents. La première était manifestement impossible et posait de probables problèmes constitutionnels. Il n'en restait qu'une : celle que vous proposez, monsieur le président

qui se sont mobilisés- des milliers et des milliers de personnes -, à Paris et dans toute la France. Je pense, madame la ministre, que cela a contribué à votre prise de conscience. Du moins, je l'espère ... Mais je déplore fortement, avec l'ensemble des membres de mon groupe, que vous n'ayez pas perçu

Nous avons abrégé la discussion. Nous avons pris le parti, d'ailleurs de manière consensuelle, non pas de cesser l'examen du PLFSS, mais de le reprendre

Il comprend des mesures nouvelles très importantes pour nos concitoyens. Un certain nombre d'articles ont été adoptés à l'unanimité par l'Assemblée nationale, car ils comprennent de très belles mesures. Nous aurons l'occasion d'en débattre. Je reviendrai sur la critique qui nous est faite de ne pas considérer le Parlement ou de ne pas entendre ses alertes. Depuis deux ans que nous nous connaissons, j'ai sans arrêt travaillé de concert avec vous. Vous m'avez alertée sur la crise des Ehpad, nous avons travaillé à un

Voilà ce que, comme tous les soignants, j'ai entendu. Ensuite, la loi HPST a réduit la part des personnels soignants dans la gouvernance hospitalière. Ces réformes successives ont désespéré l'hôpital public. Nous devons maintenant prendre en compte cette désespérance et

Il considère que l'hôpital public est un investissement pour notre société. Il l'a redit publiquement aux soignants aujourd'hui. Je pense qu'il était très important qu'il s'exprime en cette période de très grande tension hospitalière.

le résultat du scrutin n° 36 : Le Sénat n'a pas adopté. La troisième partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 n'ayant pas été adoptée, la quatrième partie est considérée comme rejetée.